? L'avis est défavorable, parce que les propositions de travaux contenues dans les audits énergétiques visent une diminution de la consommation d'énergie finale des logements rénovés. La réduction de la consommation d'énergie conduit déjà à une baisse

Pour les logements de catégorie E, F et G, l'audit énergétique comprendra des propositions de travaux par étape. La première étape de ce parcours permettra au minimum d'atteindre la classe E.

Mme la rapporteure rejeté. Je vous rappelle que l'objectif est d'abord de lutter contre les passoires énergétiques, qui sont des logements de catégorie F ou G, dont la mise en location sera interdite à compter de 2028. C'est pourquoi la première étape est d'atteindre la classe E. Dans un second temps, l'objectif est d'atteindre une rénovation performante ou globale, soit la classe B. L'avis est donc défavorable.

des dispositions réglementaires relatives à la qualité de l'air, ce qui me paraît être une très bonne idée pour éviter l'attentisme du Gouvernement sur ce sujet

qui engage sa responsabilité et relève d'un statut propre et réglementé. La réalisation de ces diagnostics entraîne un surcoût important pour les organismes HLM. C'est pourquoi l'amendement n° 1600 vise à autoriser les organismes HLM qui disposent des compétences nécessaires pour effectuer ces diagnostics à les faire réaliser en interne.

l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Ce dispositif pourra être suivi et évalué jusqu'en 2030. À compter de cette date, il est proposé de mettre en place un levier supplémentaire pour éradiquer les logements qualifiés de passoires thermiques pour être mis en vente, les logements relevant des catégories E, F et G devront faire l'objet d'une rénovation performante soit par le propriétaire, soit par l'acquéreur. Cette proposition permet de définir une trajectoire d'obligation de rénovation cohérente, qui s'échelonnera dans le temps

de la rénovation énergétique des logements, l'articulation du dispositif proposé avec l'interdiction de louer des logements classés F et G à compter du 1 janvier 2028 soulève plusieurs questions. En effet, cette interdiction, qui se cumule, je vous le rappelle, un éventuel conditionnement de la vente de ces logements à compter du 1 janvier 2030, risque de pénaliser très lourdement les propriétaires qui ne pourront plus louer leur logement

Les mesures incitatives mises en place depuis des années sont insuffisantes en termes de nombres de rénovations réalisées par an et de qualité. Elles ne nous permettent pas de remplir nos objectifs climatiques.

ainsi proposé de mettre en place un service d'accompagnement des ménages soumis à cette obligation par un tiers de confiance. Il s'agit là d'un compromis constructif entre une obligation dure et la simple incitation proposée par le Gouvernement. Il résulte d'une très large coalition d'acteurs : industriels, financiers, syndicats, réseaux de collectivités, ONG et associations de consommateurs. Surtout, il s'agit là d'une occasion historique de faire de la France la championne de la rénovation énergétique performante des logements. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Le moment est venu de changer d'échelle : pour le climat, pour la justice sociale, ne repoussons pas cette décision. Très bien ! Quel est l'avis de la commission

Toutefois, mon cher collègue, en voulant imposer une obligation conditionnelle de rénovation performante des logements à compter du 1 janvier 2024 lors de la vente, vous méconnaissez les apports d'une rénovation énergétique progressive par gestes et, de fait, les contraintes financières

l'avis du Gouvernement ? préconise le rapport Sichel, qui a été intégré dans ce projet de loi. En matière d'obligations, nous avons choisi de rendre impossible la mise en location des passoires thermiques et donc de différencier la situation des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants.

Madame la rapporteure, pour inciter les propriétaires bailleurs de passoires thermiques à accélérer leur rénovation, il faut qu'il soit moins rentable pour eux de louer leur bien qu'un logement conforme aux normes environnementales. À cet égard, il me semble que l'incitation la plus efficace-

En cas de contestation, il appartiendra au bailleur de démontrer que son logement ne relève pas de ces catégories. Nous proposons par ailleurs de supprimer le délai de trois mois pour contester ce complément de loyer. Ce délai, trop contraint pour les locataires, n'est pas justifié. La parole

celle de la rénovation et celle du coût de l'accès au logement. L'encadrement des loyers a pour vocation non pas d'encourager les bailleurs et les propriétaires à rénover leur logement, mais bien de lutter contre le logement cher et donc contre l'exclusion du marché du logement locatif d'un trop grand nombre de nos concitoyens, alors que l'offre de logements abordables n'est pas suffisante. Nous craignons ainsi qu'exclure les logements rénovés de l'expérimentation ne conduise à un renchérissement du niveau des loyers, dans un contexte où ceux-ci restent particulièrement élevés. Nous considérons pour notre part, alors que nous affrontons une crise sociale sans précédent, alors que notre pays compte un million de pauvres supplémentaires et que le taux de chômage va prochainement atteindre un pic, qu'il n'est pas opportun d'aller en ce sens et d'exclure nos concitoyens les plus fragiles de l'accès au logement en renforçant le décalage entre les capacités contributives des ménages et le niveau des loyers. Nous proposons donc la suppression de cette disposition. l'amendement n° 1131. La commission a adopté une disposition prévoyant que, en cas de travaux relevant de la rénovation performante réalisés sur des logements classés F et G par un propriétaire bailleur, le loyer puisse ne plus être encadré. Les travaux de rénovation ne justifient pas la fin de l'encadrement des loyers, bien au contraire. Nous sommes opposés à toute dérogation dans le cadre de l'expérimentation en vigueur parce qu'elle fragiliserait forcément le dispositif et parce que le locataire n'a pas à porter cet effort financier,

de l'article, qui exclut l'application du deuxième alinéa de l'article 140 de la loi ÉLAN, lequel prévoit justement un complément éventuel de loyer là où les loyers sont encadrés.

du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

Varaillas, sur l'article. L'article 42 est présenté comme l'une des mesures phares du projet de loi, car il prévoit l'interdiction de location des passoires énergétiques.

avant d'engager des recours qui pourraient, au surplus, les priver de leurs APL. En commission, nous avions d'abord pensé revenir sur les échéances, afin de les rapprocher, mais cela ne changerait rien non plus. Faute de sanction, faute d'appui aux locataires leur permettant de faire respecter leurs droits, cet article restera lettre morte.

pour tous les propriétaires, occupants et bailleurs, copropriétés, bailleurs sociaux et maisons individuelles. Elle prévoyait également des mécanismes de sanction, malheureusement absents du présent projet de loi. Tant que l'interdiction nécessitera une décision judiciaire, elle sera inefficace, car les services de l'État et les magistrats n'ont malheureusement ni le temps ni les moyens d'effectuer les vérifications nécessaires.

À défaut, et c'est inédit en droit français, l'article 42 prévoit une interdiction pure et simple de mise en location. Cet article permettra ainsi de lutter contre ces logements particulièrement énergivores, d'où l'énergie s'échappe à travers les murs, les portes, les fenêtres et les toits, provoquant des émissions de gaz à effet de serre. Il crée également un véritable mécanisme de protection des locataires, lesquels sont d'ailleurs les premières victimes de la précarité énergétique.

leur responsabilité pourra être engagée par leurs locataires, d'abord au travers d'un mécanisme de conciliation. En l'absence d'accord, le juge interviendra et pourra mettre les propriétaires en demeure de réaliser les travaux et de remettre le logement aux normes.

de société anonyme HLM au groupe Maisons & Cités, de nombreux travaux de rénovation à long terme sont entrepris pour assurer la préservation de ce patrimoine, en grande partie classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Le parc de logements des cités minières est encore occupé à 28 % par des ayants droit de mineurs. Le groupe Maisons & Cités assure la gestion de ce parc, composé de 63 000 logements répartis sur l'ensemble de l'ex-bassin minier.

de vue thermique, les prescriptions imposées sont cohérentes avec les ambitions mises en avant par le Gouvernement dans les textes qui sont actuellement en discussion. Toutefois, la rénovation de ce parc

Il convient de rappeler ici que ce patrimoine n'était pas jusqu'à présent soumis à DPE, puisqu'il est antérieur à 1948. Compte tenu du statut et des particularités de ce parc historique,

? Il me semble, mes chers collègues, que ces amendements sont satisfaits, car la commission a d'ores et déjà prévu, à la demande de la commission de la culture, des exceptions architecturales, patrimoniales, techniques et financières, lorsque les coûts des travaux sont disproportionnés par rapport au calendrier d'interdit de location. Les conditions de ces exceptions seront précisées par un décret en Conseil d'État, comme le prévoit l'article 39 que nous avons voté.

L'engagement financier de l'État est important : plus de 10 millions d'euros par an depuis 2018, et ce pour une durée totale de dix ans, dans le cadre de l'Engagement pour le renouveau du bassin minier, que vous avez cité.

Il est donc raisonnable d'espérer qu'aucun de ces logements ne tombera sous le coup du critère de décence. Par ailleurs, il me paraît difficile d'envisager une exception à ce critère pour ces seuls logements, car cet intérêt architectural ou patrimonial particulier n'est pas un motif valable de dérogations, au-delà des dérogations que Mme la rapporteure pour avis a déjà citées. Parce que nous saurons, de toute façon, atteindre notre objectif, et parce que l'exception prévue est générale, je demande le retrait de ces deux amendements.

Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 6,6 millions de nos concitoyens vivent dans une situation de précarité énergétique et 12 millions de personnes ont froid chez elles ou dépensent trop d'argent pour se chauffer.

pensez-vous sincèrement que beaucoup de locataires engageront des démarches juridiques, chronophages et coûteuses, sachant en outre que les locataires des logements les plus indécents ou les plus insalubres sont aussi, on le sait, Dans les zones où le marché est tendu, les locataires ne veulent pas prendre le risque de perdre leur logement et ils hésitent donc souvent à faire respecter leurs droits en s'attaquant à leur bailleur. C'est pourquoi nous proposons de garantir une réelle interdiction de nouvelles mises en location de logements considérés comme des passoires thermiques,

L'atteinte du niveau BBC pour l'ensemble du parc résidentiel en 2050 semble donc impossible si le rythme et la qualité actuels des rénovations restent inchangés. » Alors qu'il faut multiplier ce rythme par dix, nous regrettons que le financement de MaPrimeRénov'soit encore inférieur au crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui était lui-même insuffisant. à l'énergie et au climat aurait pu constituer l'occasion de prévoir l'interdiction progressive de la location des logements les plus énergivores, conformément au programme présidentiel de 2017 qui, je le rappelle, préconisait la rénovation de la moitié des passoires énergétiques dès 2022 et l'interdiction de leur location à compter de 2025. Certes, cela méritait un accompagnement des propriétaires, qui a tardé à se concrétiser. Nous regrettons, en outre, la suppression de l'audit énergétique pour la location des logements F et G, alors que le changement de titulaire du bail constitue le meilleur moment pour réaliser des travaux de rénovation. Notre amendement vise donc à avancer de trois ans les dates à partir desquelles les logements les plus énergivores seront considérés comme indécents, afin d'accélérer la dynamique de rénovation du parc de logements

est à Mme Viviane Artigalas. Cet amendement a pour objet de faciliter la compréhension des dispositions liées au niveau de performance énergétique, afin de lever toute incertitude sur le périmètre et les dates d'application des nouvelles mesures relatives à la décence du logement.

Nous souhaitons que soit interdite plus rapidement la location de ce type de logements et que l'échéancier de la transition soit plus resserré dans le temps. La date de 2040 nous semble beaucoup trop lointaine. Cette trajectoire nous éloignera encore davantage de nos objectifs de réduire de

En 2048, nous en serons à la vingt et unième législature et la plupart d'entre nous ne sera plus de ce monde. J'aimerais éviter de voter une loi dont je ne suis pas certain de voir l'application de mon vivant. Certes, gouverner c'est prévoir, mais restons dans les limites d'une génération ! Il est absurde de se projeter dans vingt-sept ans. Mes chers collègues, si nous ne sommes pas capables de rénover le parc de logements classés D d'ici à 2040, je doute de notre capacité à enrayer le réchauffement climatique en deçà de 4 degrés !

contre son propriétaire et exiger qu'il effectue des travaux d'isolation. Mais, en pratique, très peu de locataires actionneront cet outil. Dans les zones où le marché est tendu, les locataires sont souvent réticents à faire respecter leurs droits en s'attaquant à leur propriétaire,

Nos amendements visant à inscrire dans la loi une sanction ayant été malheureusement rejetés, nous renvoyons à un décret le soin de fixer ces sanctions, laissant ainsi le temps au Gouvernement de procéder

proposons que ce décret soit pris avant le 1 janvier 2025, date à laquelle les propriétaires de passoires thermiques classées G seront tenus, au titre du présent article 42, de réaliser des travaux de rénovation énergétique s'ils souhaitent louer leur logement. Il s'agit donc d'une date butoir. Quel

de travaux. Il s'agit de la meilleure manière de rendre effectives les obligations et l'éradication concrète des passoires thermiques aux horizons fixés dans le présent article. Sans sanction à caractère dissuasif, nous craignons que les obligations prévues ne restent lettre morte. La rédaction que nous proposons vise ainsi à clarifier le caractère d'ordre public des obligations définies et des sanctions concomitantes aux obligations de travaux, posées par l'article 20-1 Il s'agit également de parfaire l'information du consommateur, qui est le pivot, avec ces dispositions, de la lutte contre la non-décence et de la résorption des passoires thermiques. Il convient notamment de sanctionner un bailleur qui ne respecterait pas le décret « décence » avant de louer, notamment en

En effet, l'intervention de la CAF ne semble pas devoir être mentionnée dans une loi qui régit les rapports entre les propriétaires et les locataires. Enfin, il paraît très difficile de combiner un bail différé et la suspension des APL ou du loyer. J'émets donc, comme en commission, un avis défavorable.

juge avait besoin d'une expertise, malgré les constats de non-décence que la CAF aura généralisés, celle-ci doit être mise à la charge du bailleur fautif. Dans ce cadre, le juge peut prononcer une réduction provisionnelle du montant du loyer de 50 % à 75 %, avec ou sans consignation. Nous proposons également que l'organisme payeur et la commune ou l'EPCI dont dépend le logement puissent s'associer à l'action du locataire, notamment par la voie d'une intervention à titre volontaire devant le juge. Avec ce nouveau dispositif, nous souhaitons rendre effectives les dispositions de cet article qui visent à rendre indécents les logements considérés comme des passoires thermiques et donner concrètement aux locataires les moyens de faire respecter leurs droits. À défaut, malgré les bonnes intentions, ces dispositions seront inopérantes.

au locataire. En cas d'appel de garantie de la copropriété, le juge ne pourra donc pas lui imposer de réaliser des travaux sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, pas plus qu'il ne pourra imposer au bailleur de réaliser des travaux qu'il ne peut, juridiquement, décider. Cet amendement mobilise de manière inopérante la procédure civile d'appel en garantie. Pour cette raison, l'avis est défavorable.

a émis 50 propositions afin d'engager la transformation écologique du système de santé. L'État doit accompagner ces investissements. Les travaux de rénovation énergétique des logements bénéficient d'un taux réduit de TVA à 5,5 %. Il s'agit, au travers de cet amendement, d'étendre l'application de ce taux réduit de TVA aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, afin d'accompagner l'amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments. Quel

l'amendement n° 186. Cet article, inséré en commission, crée le risque d'une augmentation des loyers des logements concernés. La mise en congé pour travaux de rénovation devrait donc être assortie d'une obligation de louer à nouveau, sans complément de loyer.

la rénovation énergétique ne doit pas se faire au détriment des locataires. Or il existe un risque réel de détournement d'un tel congé pour rénovation énergétique lorsque le bailleur souhaite libérer le logement. Par ailleurs, en l'état du droit, le fait que le bailleur souhaite réaliser des travaux constitue déjà un motif légitime et sérieux de congé, sous réserve que la réalisation de ces travaux nécessite le départ du locataire. La jurisprudence encadre donc déjà suffisamment l'hypothèse de travaux de rénovation énergétique. Pour ces raisons, j'émets un avis favorable sur ces amendements de suppression.

Varaillas. Par cet amendement, nous souhaitons affirmer le rôle des collectivités en soutien des locataires. Nous proposons donc l'instauration d'un arrêté de précarité énergétique. Ainsi, le maire pourrait, en vertu de cet arrêté, prescrire l'exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d'habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1 janvier 2028 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont le niveau de performance énergétique et climatique relève de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d'énergie excessive. permettre au maire de faire procéder à tous contrôles qui lui paraissent utiles à l'effet de vérifier la performance énergétique du logement. Cet arrêté de précarité énergétique s'intègre ainsi dans les pouvoirs et procédures des polices bâtimentaires, décrites par les articles L. 511-1 à L. 511-22. En complément, nous prévoyons que, si ces mesures engagent un besoin d'hébergement provisoire, alors le droit à réintégration dans le logement rénové est acquis. Nous considérons que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir sur cet enjeu essentiel, en complément et en soutien des locataires, qui ne sauraient être les seuls à agir. Quel est l'avis de la commission

communs défectueux, des matières dangereuses et le préfet des autres aspects. Enfin, le maire ne peut pas procéder à des contrôles sans condition. L'article L. 152-13 du code de la construction et de l'habitation, prévoit : « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire

ne se limite pas à l'amélioration de la performance énergétique, mais inclut également celle de la performance climatique. Par ailleurs, il est proposé de rappeler explicitement la priorité donnée aux rénovations performantes au 17° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, il paraît opportun de rappeler que les recommandations ne doivent pas porter sur des travaux ayant pour conséquence un accroissement des émissions de gaz à effet de serre.

à établir une distinction claire entre les missions d'information et de conseil offertes à tous les ménages par le service public de la performance énergétique de l'habitat et l'accompagnement, lequel sera obligatoire pour obtenir certaines aides publiques. Les organismes qui tiennent les guichets, ainsi que les collectivités, pourront aussi assurer la mission d'accompagnement, s'ils le souhaitent et s'ils disposent des compétences requises. L'amendement vise également à préciser que les situations dans lesquelles l'accompagnement sera obligatoire pour bénéficier des aides ne devront pas être limitées aux rénovations performantes et globales. Elles devront également inclure d'autres cas de figure qui mobilisent un montant important d'aides publiques afin de s'assurer que les travaux envisagés sont bien adaptés et suffisamment ambitieux. Il tend à préciser que le financement pourra s'adosser aux certificats d'économies d'énergie et à prévoir une simplification des modalités de reconnaissance des opérateurs d'accompagnement. Ceux-ci sont des acteurs clés pour massifier l'offre et devront être opérationnels sur l'ensemble du territoire dès le 1 janvier 2023, voire avant. Or, comme nous l'avons expérimenté, la montée en puissance des mécanismes d'aide et de conseil est parfois plus lente que l'engouement des Français pour ces travaux, ce qui peut générer des temps d'attente et des insatisfactions.

de sélection permettrait néanmoins de conserver une exigence forte concernant les garanties de compétences et de probité. Un décret prévu en Conseil d'État y veillera. Mme Viviane Artigalas. L'article 43 prévoit que les guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique déployés sur l'ensemble du territoire peuvent « assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement. » Notre amendement vise à compléter cette mission en y intégrant l'identification des ménages en situation de précarité énergétique.

Dans l'objectif de massification des rénovations énergétiques, il est essentiel que le service public de la performance énergétique de l'habitat oriente prioritairement les ménages vers des rénovations performantes et les accompagne dans leur parcours de rénovation, en levant les freins identifiés.

présente encore des risques quant à la neutralité du conseil apporté aux particuliers. Cet amendement vise à permettre que la mission d'accompagnement remette aux particuliers une liste de professionnels locaux en fonction des travaux envisagés et ne procède pas à une sélection de professionnels, comme cela est envisagé dans le texte, le choix de l'entreprise appartenant au client. De même, le coût des travaux peut évoluer en fonction des précisions apportées par les professionnels et de l'état du bâti et ne peut donc être fourni que de manière indicative ou estimative par l'opérateur. Enfin, le seuil proposé de 5 000 euros de travaux pour bénéficier d'une mission d'accompagnement paraît inadapté. En effet, ce montant correspond le plus souvent à un seul geste,

aux opérations d'autoconsommation collective, afin de valoriser non seulement la baisse de la consommation globale d'énergie, mais également la lutte contre la précarité énergétique permise par ces opérations. Cette bonification reprendra le même schéma que celui qui a été mis en place pour le contrat de performance énergétique (CPE) et sera cumulable avec les autres bonifications. En permettant une part de consommation renouvelable à un coût moindre, les fonds privés issus de C2E viendraient ici répondre au double objectif qui leur est assigné : réduire la consommation d'énergie du réseau tout en participant à lutter contre la précarité énergétique. Cette solution de financement privé des opérations d'autoconsommation collective, qui s'inscrit dans une logique de lutte contre la précarité énergétique pour les habitants d'immeubles collectifs qui n'ont pas accès à l'autoconsommation individuelle, permettra de multiplier les opérations montées notamment par les bailleurs sociaux au bénéfice de leurs locataires, sans subvention publique. Les

doivent pouvoir être réalisés soit en une seule fois par un ensemble d'entreprises, soit par étapes dans le cadre d'un parcours de travaux. L'amendement tend par ailleurs à prévoir que soient fixées les compétences exigées des opérateurs, notamment pour être à jour de l'évolution des réglementations en

tend ainsi à respecter l'esprit des travaux de la commission des affaires économiques, qui a eu à coeur de prévoir un reste à charge moindre pour les ménages.

avec le reste de la législation. Il y est ainsi fait référence à la performance climatique, qui n'existe pas au sens du DPE, même si celui-ci intègre naturellement les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, en posant le principe selon lequel les travaux de rénovation énergétique ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, à reprendre un principe existant pour les certificats d'économies d'énergie à l'article L. 221-7-1 du code de l'énergie ou qui est prévu pour toutes les autres opérations à l'article 46 du

d'abord, il tend à supprimer la procédure d'agrément des accompagnateurs et, partant, tout le cadrage intégré à cet article par notre commission : l'exigence d'une indépendance et d'une impartialité, la possibilité pour les collectivités territoriales,

des évolutions surprenantes, comme la suppression de la mission d'accompagnement des guichets et de la fonction de rédacteur des notaires ou encore l'ajout d'une mission d'information sur le bruit, laquelle, aussi utile soit-elle,

pour les ménages modestes, puisque la commission des affaires économiques a prévu leur financement les certificats d'économies d'énergie. Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont mentionnés parmi les acteurs vers lesquels les guichets peuvent orienter les consommateurs. Les copropriétaires ne sont pas exclus du service public de la performance énergétique et de l'habitat, puisque l'article fait bien référence aux consommateurs d'énergie, sans exclusive. Enfin, la mission d'accompagnement prévoit des garanties et des compétences pour la sélection des accompagnateurs Sichel.

rectifié et 1597 rectifié : l'article prévoit déjà des exigences en matière de qualification et de compétences, notamment sur les plans technique, architectural et patrimonial. Par ailleurs, le relèvement du seuil de la conditionnalité des aides de 5 000 à 15 000 euros écart considérable par rapport à la mission Sichel, à laquelle notre commission a entendu se référer. Ensuite, l'attribution au service public de la performance énergétique de l'habitat d'une mission de suivi de la précarité énergétique me semble être satisfaite, puisqu'une telle mission est actuellement menée par l'Observatoire national de la précarité énergétique par sa trentaine d'organismes partenaires. Enfin, l'amendement n° 60 rectifié tend à prévoir une concertation préalable des professionnels pour l'élaboration du décret.

tend à créer une nouvelle mission d'identification des ménages en situation de précarité énergétique, mais, comme l'a dit Mme la rapporteure pour avis, cette mission est déjà couverte par de nombreuses instances, dont l'Observatoire national de la précarité énergétique. L'avis est donc défavorable.

qui vise à rendre l'accompagnement gratuit pour les ménages les plus modestes. Tout l'objet de l'action du Gouvernement est de bien différencier et de limiter le reste à charge pour les ménages les plus modestes.

est à Mme Annick Billon. Cet amendement, déposé par notre collègue Jean-Michel Arnaud, a pour objet d'orienter les ménages vers un interlocuteur en capacité d'apporter des solutions techniques personnalisées.

Il s'agit ainsi de consolider le rôle de la mission d'accompagnement telle qu'il résulte des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat.

De plus, cela décalerait l'entrée en vigueur des autres dispositions du texte qui, en l'absence d'un tel délai, seraient d'application immédiate, à compter de la promulgation de la loi- il en va notamment ainsi des nouvelles missions

En complémentarité avec d'autres organismes, elles exercent de nombreuses missions en faveur de la transition énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, elles accompagnent l'élaboration des schémas et des plans territoriaux et apportent un soutien en ingénierie territoriale aux particuliers et aux collectivités territoriales.

Après une reconnaissance législative tardive, en 2015, leur statut juridique et fiscal demeure fragile, comme en témoignent les nombreuses questions parlementaires déposées à cet égard. Sans une prise de position claire de l'administration fiscale, il est à craindre qu'une partie de leurs prestations ne soit considérée comme relevant du domaine concurrentiel. ce cas, elles seraient soumises aux impôts commerciaux, ce qui les exposerait à un risque de rattrapage fiscal sur plusieurs années. Pourtant, les ALEC n'entendent pas se substituer au secteur concurrentiel. Il est donc nécessaire que le Gouvernement clarifie leur statut, afin de lever cette incertitude, qui risque de peser sur leur fonctionnement, alors que leur travail est essentiel en matière de climat et de transition énergétique. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi l'étendue des missions actuelles

favoriser la production d'énergie renouvelable locale, de gagner en autonomie énergétique et de lutter contre la précarisation des habitants et des acteurs économiques. Leur action vise enfin à limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine. La parole

réparties sur l'ensemble du territoire national. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail remarquable qu'elles accomplissent localement pour favoriser la mise en oeuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en informant, en sensibilisant, en conseillant, de manière indépendante et objective, les citoyens, ainsi que les acteurs publics et privés.

et de la relance à cet effet. Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable sur cette série d'amendements.

sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ?

de la performance énergétique et visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments d'habitation classés F ou G. Il s'agit de mettre en place une incitation plus forte aux rénovations performantes. En effet, le gain obtenu par le passage d'une classe F ou G à une classe E paraît trop faible pour permettre d'atteindre les objectifs fixés à grande échelle. Il est donc nécessaire d'encourager plus vigoureusement la rénovation performante de ce type de logements. Les rénovations globales, dont la définition s'approche de celle de la rénovation performante, ne représenteraient à ce jour que 0,2 % des travaux de rénovation, alors même qu'elles doivent être mises en oeuvre à grande échelle pour permettre d'atteindre les objectifs fixés.

Quel est l'avis de la commission la rédaction proposée établit un principe très large, qui s'appliquerait ainsi à l'ensemble des dispositifs budgétaires ou fiscaux de soutien à la rénovation énergétique, dont l'objet, le public

Enfin, et surtout, s'il était adopté, cet amendement contreviendrait aux travaux de la commission des affaires économiques, qui a souhaité que la nouvelle définition de la rénovation énergétique performante n'induise pas d'effet de bord négatif sur les dispositifs budgétaires ou fiscaux en direction des ménages.

tous les travaux améliorant la performance ou seulement ceux qui font changer de classification ? Dès lors qu'il y a amélioration de la performance, les travaux méritent d'être inscrits

Cependant, la mobilisation de ce fonds ne signifie pas pour autant délivrance de prêts aux ménages les plus modestes, lesquels en ont pourtant besoin pour financer le reste à charge de leurs travaux.

destinés aux ménages modestes et très modestes, ont été délivrés en 2020, soit moins de 1 % des éco-PTZ. Cet amendement a donc pour objet de fixer, dans la convention qui permet aux banques de bénéficier de la garantie du FGRE, des objectifs de délivrance des éco-PTZ et des prêts avance mutation garantis. Ces objectifs permettront d'améliorer la distribution des prêts dédiés à la rénovation énergétique auprès des ménages modestes et ainsi d'éviter les renoncements aux travaux, faute de solution bancaire. Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique pourra enfin jouer pleinement son rôle, notamment social, en accomplissant les missions qui lui sont assignées.

la garantie du fonds à l'éco-PTZ consenti sans condition de ressources. Or tel n'est pas son objectif. J'émets donc un avis défavorable

Dans un contexte où le programme Action coeur de ville et le plan Logement d'abord ont pour objectif un recentrage de l'intervention des propriétaires bailleurs, et où les crédits de la ligne budgétaire unique (LBU) se trouvent désormais réduits, nous constatons un émiettement des capacités de financement public des politiques publiques du logement outre-mer.

défavorable. Quant aux deux autres amendements, l'avis est également défavorable. En effet, l'intégration d'une nouvelle association d'élus au sein du conseil d'administration aurait pour conséquence de nommer 12 nouvelles personnes- 6 membres titulaires et 6 membres suppléants afin de respecter les contraintes légales d'équité entre les trois collèges du conseil d'administration de l'ANAH. Or je vous rappelle que ce conseil est déjà composé de 24 membres titulaires et de 24 membres suppléants, ce qui est largement suffisant.

que l'un des deux soit issu d'un territoire ultramarin. Néanmoins, je voudrais vous rassurer sur le fait que l'ANAH et le ministère du logement prennent en compte la spécificité des situations ultramarines. Dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022, la conférence du logement en outre-mer a permis de conclure au maintien d'un engagement fort de l'État sur le sujet. En ce qui concerne l'ANAH, une convention pluriannuelle d'objectifs et de partenariat entre l'agence, le ministère des outre-mer et le ministère chargé du logement, a été signée, il y a à peine quelques semaines.

Cuypers. Cet amendement vise à étendre le champ des actions relevant du projet pluriannuel de travaux aux actions conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. un urbanisme rénové (ALUR) la réalisation des installations permettant aux occupants et à leurs visiteurs de recourir à des modes de transport à très faibles émissions, notamment les emplacements pour vélos, les installations de recharge de véhicules électriques ou de véhicules à hydrogène sur les emplacements de stationnement, y compris ceux réservés aux visiteurs. ceux réservés aux visiteurs. De plus, il est spécifié que le plan ne peut avoir pour effet d'accroître les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le cas où un changement d'énergie serait envisagé.

De mon côté, l'avis est défavorable pour deux raisons. La première tient à ce que cet amendement vise en particulier le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques au sein des immeubles d'habitation.

être source de désordres et de prises de responsabilité non maîtrisées. La densification par agrandissement, la surélévation et l'amélioration des caractéristiques de l'enveloppe bâtie du fonds servant pourrait être compromise, rendant obsolètes les dispositions vertueuses de la loi à son égard. La parole est à

M. Martin Lévrier. L'article 44 vise à faciliter les isolations thermiques en permettant au propriétaire du mur d'un bâtiment existant de procéder à son isolation par l'extérieur, en application d'un droit de surplomb sur la propriété voisine. Jusqu'à présent, si les matériaux d'isolation empiétaient sur le terrain d'à côté, un accord du voisin était nécessaire, faute de quoi l'isolement devait se faire par l'intérieur. Cet article transcrit pleinement l'objectif de ce projet de loi : lutter contre le dérèglement climatique par l'accompagnement très concret des Français dans leur quotidien.

En effet, les aides proposées par l'État, qui mobilisent un budget de plus en plus considérable pour remplir les obligations liées à la stratégie nationale bas-carbone, ne doivent pas finir dans les poches d'acteurs frauduleux qui rejoignent le marché uniquement pour escroquer les ménages. Qui n'a pas entendu parler des rénovations à un euro qui ont ruiné certains ménages autour de nous ? Les pouvoirs publics doivent protéger nos concitoyens. Nous demandons donc que soit effectué, sous la responsabilité de l'État, et au travers de bureaux indépendants et certifiés, un contrôle des chantiers. garantira que les aides mises en place permettent une rénovation énergétique efficace, effectuée par des professionnels fiables. Je précise que la charge de cette mesure doit être assumée par l'entreprise.

d'élargir cette exception aux logements mis en location, plus particulièrement ceux qui sont loués pour un prix modeste. Tel est l'objet de cet amendement. Quel Mme la rapporteure. la commission a adopté des dispositifs incitatifs à l'égard des bailleurs pour mieux les accompagner encore dans leur démarche de rénovation énergétique. Enfin, le seuil qui est mentionné dans votre amendement est très élevé. Il s'agit de passoires thermiques et il convient de privilégier la protection des locataires. Je pense, néanmoins, que votre amendement est satisfait. Je vous demande donc de le retirer

un logement qui est classé F sera déclaré indécent. Le locataire pourra ainsi exiger sa mise aux normes et obtenir une réduction provisoire du loyer. Ce mécanisme vient sanctionner le non-respect d'obligations antérieures. Il me semble donc logique

ou tous travaux de rénovation énergétique. Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement. Celle-ci ne peut être réalisée que par des opérateurs agréés par l'État ou l'ANAH. À ce titre, les OPH doivent pouvoir être agréés en qualité d'opérateurs chargés de la mission d'accompagnement définie au nouvel article L. 232-3 du code de l'énergie, dans le cadre du service public de la performance énergétique, l'appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétique, et l'assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.

Comme la commission l'a déjà fait pour les offices publics de l'habitat, ces amendements visent à étendre aux entreprises sociales de l'habitat (ESH) la possibilité de réaliser pour le compte de tiers, des travaux de rénovation énergétique. En revanche, il ne me paraît pas nécessaire de prévoir leur agrément comme accompagnateurs des ménages au titre du service public de la performance énergétique de l'habitat, car rien ne l'empêche à ce stade. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de l'amendement n° 540 rectifié,

l'avis du Gouvernement ? Cet amendement vise à compléter la rédaction adoptée en commission sur l'extension des compétences facultatives des OPH à la réalisation pour le compte de tiers de toutes opérations ou tous travaux de rénovation énergétique. Autant je suis favorable à l'accompagnement ciblé dans des copropriétés mixtes, autant il me semble

de l'aménagement et du numérique (ÉLAN), en matière d'opération de construction et d'aménagement que ces sociétés peuvent effectuer pour le compte de ces personnes publiques. Un tel élargissement de leurs compétences permettrait, également, de mieux garantir le respect des objectifs fixés par cette loi en matière de réduction de l'empreinte carbone des logements. D'autres personnes morales de droit public se trouvent, par ailleurs, associées de ces sociétés, notamment les établissements publics de coopération intercommunale qui sont intéressés par cette capacité d'intervention. L'amendement vise donc à les intégrer parmi les bénéficiaires potentiels.

Les coopératives d'HLM ont développé une expertise reconnue en matière de réhabilitation énergétique, tant dans le domaine de l'ingénierie technique que dans celui Présentes de manière pérenne sur des territoires tendus comme détendus, elles sont des interlocuteurs de confiance, notamment pour les collectivités territoriales et les copropriétés qui seront en première ligne pour activer, voire piloter, cette dynamique de massification. C'est pourquoi le présent amendement vise à donner la capacité aux coopératives d'HLM d'agir comme tiers de confiance et ensemblier au service de la dynamique de massification, laquelle inclut tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publiques ou privées. À ce titre, les coopératives d'HLM doivent pouvoir être agréées en qualité d'opérateur chargé de la mission d'accompagnement définie au nouvel article L. du code de l'énergie, dans le cadre du service public de la performance énergétique, pour appuyer la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques, et assurer l'assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cet amendement vise en outre à garantir une cohérence dans les compétences des organismes d'HLM. En effet, le texte du projet de loi issu des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable accorde déjà cette capacité aux OPH.

plus petite, mais qui n'est assurément pas la moins sociale, tant s'en faut ! Elle contribue, par son essence même, à l'effort en matière de logement. Elle a notamment fait beaucoup pour l'accession sociale à la propriété,

consomme obligatoirement une part minimale de gaz renouvelable son offre d'énergie. Grâce à l'excellence énergétique des nouveaux bâtiments, le consommateur ne verra pas sa facture s'emballer et les coûts de construction demeureront contenus par l'absence de normes supplémentaires de production. Cette obligation nouvelle sera mentionnée dans les contrats de location, les actes de vente et les règlements de copropriété. L'information de l'occupant sera donc certaine. Le propriétaire conservera une liberté de choix dans l'énergie, mais s'il choisit le gaz comme énergie de chauffage, celui-ci devra être renouvelable. L'information préalable du locataire lui permettra de faire un choix éclairé, tant sur le logement que sur son fournisseur de gaz vert. Le locataire disposera ainsi, et malgré une nouvelle obligation, d'une plus grande liberté et d'une plus grande information que pour les logements raccordés aux réseaux de chaleur urbains. La numérotation des articles prend en compte l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I du code de la construction et de l'habitation qui entrera en vigueur au 1 juillet 2021. Quel ? Si le gaz renouvelable doit être promu pour diversifier notre mix énergétique, le dispositif que vous proposez pourrait se révéler inefficace. D'une part, le recours à une évolution législative n'est pas utile, puisque le travail en cours sur le dispositif Méthaneuf, engagé par la filière et par le Gouvernement, peut lui être préféré. D'autre part, les sites de production de biogaz n'existent pas sur l'ensemble du territoire, de sorte qu'une obligation uniforme pourrait être

Alors que le plan de relance devrait permettre une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est primordial d'intégrer les enjeux liés à l'économie circulaire

Billon. Les certificats d'économies d'énergie constituent l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Aussi, cet amendement vise à accroître le contrôle du Parlement sur les C2E en prévoyant que, avant chaque nouvelle période, le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de ce dispositif sur la période s'achevant, notamment les économies d'énergie réalisées au regard de son coût pour les entreprises obligées, les effets sur le prix de l'énergie pour les consommateurs

Elle a prévu qu'ils évoluent selon une fourchette fixée par le Parlement dans le cadre de la loi quinquennale. En outre, elle a posé le principe d'une évaluation par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des gisements d'économies exploitables.

Cela poserait un problème de concurrence entre les différents fournisseurs d'électricité qui ne seraient pas soumis aux mêmes obligations. Si les spécificités des ELD devaient être prises en compte, elles pourraient l'être par voie réglementaire. Ce sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, faute

C2E. Actuellement, les C2E sont imposés immédiatement sur l'exercice comptable au cours duquel ils ont été acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui affecte la trésorerie des entreprises investissant pour réduire leur consommation énergétique. Il serait contre-productif d'aider les entreprises à financer ces installations économes

Appliquer ce régime aux C2E introduirait une confusion quant à leur nature juridique : il ne s'agit pas de subventions relevant du budget de l'État, mais d'un mécanisme extrabudgétaire par

Quel est l'avis de la commission

qui concerne déjà de nombreux autres combustibles. En effet, l'utilisation d'un bois de qualité permet de réduire très fortement les émissions de CO2. Le code de bonnes pratiques pour l'utilisation des combustibles solides et indique que l'utilisation de bois ayant un taux d'humidité de 20 % peut réduire les émissions de particules de 75 % par rapport à celle d'un bois présentant un taux d'humidité de 30 %.

à M. Ronan Dantec. Par cet amendement, nous reprenons la proposition SL2.3 de la Convention citoyenne pour le climat intitulée : « Inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les espaces publics et ceux ouverts au public, ainsi que les bâtiments tertiaires

Quel est l'avis de la commission

ne peuvent pas subventionner des opérations conduisant à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du présent projet de loi, notre commission a voté l'extension de ce principe à toute opération d'économies d'énergie. Il s'agit d'appliquer ces nouvelles dispositions, de les évaluer